d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à M. Bruno Sido, auteur de alimentaire. Madame la ministre, j’appelle votre attention sur la recrudescence des attaques de loups dans le département de la Haute Marne.

Les attaques se multiplient à un rythme alarmant. Les loups prolifèrent sans contrôle. Sans prédateur naturel, la pression sur les troupeaux ne cesse d’augmenter. Les conséquences sont catastrophiques : les ovins sont stressés, l’agnelage est menacé et la filière est en grand danger. Les éleveurs n’en peuvent plus. Excédés, désespérés, ils assistent impuissants à ces attaques répétées et font face à une administration qui reste sourde à leur détresse. Certains, à bout de forces, vont jusqu’à vendre leurs troupeaux. Les moyens de protection engagés par l’État se révèlent largement insuffisants : les filets de protection, censés dissuader les loups, sont contournés ; les chiens de protection et les tirs de défense, très encadrés, ne suffisent pas. Les loups attaquent toujours. Ce n’est plus tenable. L’avenir de l’élevage ovin dans le département est en péril. Les agriculteurs veulent simplement pouvoir vivre de leur travail et exercer leur métier dans des conditions sereines. Aussi, madame la ministre, quels moyens concrets l’État compte t il mettre en place ? Quels engagements budgétaires et quelles actions durables le Gouvernement envisage t il pour protéger la filière ovine en Haute Marne ?

la prédation du loup est un sujet très difficile et je connais le désarroi de nos éleveurs. Élue moi même d’un territoire très touché, je suis résolue à agir de manière déterminée en la matière. Tout d’abord, je rappelle l’adoption du nouveau plan national d’action loup, qui, pour la première fois, une réelle ambition de protection des activités d’élevage aujourd’hui menacées. Les chiffres sont terribles : la prédation lupine, c’est plus de 4 000 constats d’attaque par an et plus de 12 000 animaux tués. Il nous faut donc réagir. En 2024, mon ministère a engagé 41 millions d’euros pour soutenir les éleveurs. Nous poursuivrons cet effort en 2025, malgré les difficultés budgétaires. En ce qui concerne les réparations, la prise en compte des dommages indirects est notre objectif. Nous avons donc anticipé une augmentation d’environ 50 % des indemnisations dans le budget 2025, pour un total de 9 millions d’euros. Pour les troupeaux non protégeables, le travail se poursuit pour faciliter la délivrance des autorisations de tirs de défense et permettre les indemnisations.

vous savez que je me suis engagée de toutes mes forces, sans tergiverser, dans le combat européen du déclassement du loup pour permettre enfin de passer d’une logique de défense à une logique de régulation de la population. Soyons clairs, monsieur le sénateur, l’indemnisation ne résout pas tout : nous souhaitons qu’il y ait moins de prédation.

Comme vous le savez, ces services jouent un rôle vital dans la surveillance sanitaire des importations animales et végétales. Ils garantissent la sécurité des consommateurs, ainsi que la protection des filières agricoles et agroalimentaires françaises. depuis plusieurs années, les professionnels du secteur signalent des dysfonctionnements notables. Ces difficultés, dues en partie à un manque d’effectifs, ont un impact sur l’efficacité des contrôles sanitaires, retardent fortement les importations et affectent la compétitivité des entreprises françaises. La situation est particulièrement catastrophique sur le port de Fos sur Mer, où des emplois locaux sont menacés. il est vital de maintenir la chaîne d’approvisionnement, tout comme le haut niveau de service, afin d’enrayer le phénomène grandissant de report des trafics vers d’autres ports européens, notamment celui de Barcelone. Face à ce constat des plus alarmants, je souhaiterais connaître les mesures concrètes que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour renforcer les moyens humains et matériels des services vétérinaires, améliorer leur fonctionnement et ainsi garantir la compétitivité des ports français. Je m’interroge également sur les perspectives

Notre objectif est bien de limiter le temps d’attente des marchandises dans les postes de contrôle frontaliers (PCF) du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (Sivep) du ministère, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité sanitaire pour les consommateurs et pour les filières agricoles et agroalimentaires de l’Union européenne. C’est dans cette perspective que, chaque année, les moyens mis à disposition de chaque poste de contrôle frontalier sont revus au regard des flux réels contrôlés

que par des vétérinaires, ce qui peut être particulièrement gênant en cas de vacance de poste. Pour éviter ces carences, un décret en Conseil d’État encadre notamment, depuis 2019, le recrutement de vétérinaires de nationalité étrangère.

En application de l’article L. 230 5 1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par l’article 24 précité, le décret du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs précise la liste des signes d’identification de la qualité et de l’origine, les fameux Siqo, et des mentions valorisantes entrant dans le décompte de l’objectif de 50 %. Il s’agit notamment des produits issus de l’agriculture biologique ou en conversion, des produits bénéficiant d’autres signes ou mentions à l’article L. 640 2 du même code, qui sont définis par décret, ou encore des produits issus du commerce équitable ou bénéficiant de l’écolabel « pêche durable ». C’est dans ce contexte que la région Bretagne soutient la mise en place du label marque « Breizhmer », avec l’ambition qu’il soit reconnu comme « Siqo Égalim mais les pouvoirs publics ne peuvent favoriser un label privé plutôt qu’un autre. En outre, ils ne peuvent autoriser les acheteurs publics à intégrer unilatéralement de nouveaux labels dans cette liste. autant, les acheteurs qui exigent des produits bénéficiant du label « pêche durable » sont dans l’obligation, conformément au code de la commande publique, de prendre également en considération les produits équivalents, c’est à dire les autres produits apportant les mêmes garanties. L’appréciation de cette équivalence est laissée au jugement de l’acheteur, lequel peut considérer qu’un faisceau d’indices existe, conformément à l’article R.

Madame la ministre, le Gouvernement prévoit il de modifier le décret du 23 avril 2019 pour reconnaître d’autres labels ? L’approche multi labels pour apprécier l’équivalence peut elle être considérée comme la procédure idoine à mettre en œuvre par les acheteurs ? Quelle position l’acheteur doit il adopter pour que cette reconnaissance soit ensuite juridiquement opposable ? La parole

Ainsi, les Siqo ne se limitent pas à un engagement ponctuel ou à la signature d’une charte. Les produits relevant de ces labels font l’objet de contrôles réguliers par des organismes de défense et de gestion pour garantir leur conformité continue au cahier des charges.

Les produits durables et de qualité entrant dans le décompte des 50 % doivent répondre à l’un des onze critères précisés à l’article L. 230 5 1 du code rural et de la pêche maritime. La volonté du Gouvernement est bien d’assurer la souveraineté alimentaire, notamment dans un objectif de soutien de l’économie agricole des territoires, de réduction de l’impact environnemental des filières et de sécurisation des approvisionnements en produits vivriers. C’est pourquoi l’utilisation combinée de certains critères permet, dans le cadre de marchés publics ou d’appels d’offres, la sélection de produits locaux, y compris hors Siqo. Ainsi, des labels privés peuvent facilement être sélectionnés. C’est notamment le cas de « Bleu Blanc Cœur ». Néanmoins, vous en conviendrez, cette liste est déjà à la fois exhaustive et souple, ce qui permet de prendre en compte certaines équivalences. Le Gouvernement n’envisage donc pas de révision des critères à ce stade. J’ajoute que

Spécialisé dans l’affinage de l’aluminium, cet acteur de l’économie locale doit pourtant surmonter des obstacles majeurs. Tout d’abord, il y a le recyclage. Bien que Sadillek contribue activement à la transformation des déchets d’aluminium, la France manque d’une politique ambitieuse avec des infrastructures adaptées pour soutenir et retenir ces déchets sur le territoire. Chaque année, nous exportons plus de 500 000 tonnes de déchets d’aluminium non traités, privant nos affineurs de matières premières pour leur activité. Cette fuite des ressources limite directement la capacité de nos industriels à augmenter leur production et contribue à notre dépendance aux importations de métal. Ensuite, il y a la compétitivité énergétique. L’affinage de l’aluminium est une activité très énergivore, avec des coûts d’énergie parmi les plus élevés en Europe. Ces charges pèsent lourdement sur les marges des entreprises et réduisent leur compétitivité, particulièrement face à des concurrents étrangers soutenus par des politiques énergétiques énergétiques avantageuses, comme en Chine. Ces difficultés conjuguées à une concurrence internationale intense et aux tensions géopolitiques mettent à mal l’ensemble de la filière aluminium française, pourtant stratégique. Avec plus de 10 000 emplois directs et un rôle clé dans des secteurs comme l’aéronautique ou l’automobile, cette filière est indispensable. Madame la ministre, quelles initiatives concrètes le Gouvernement entend il prendre pour garantir la compétitivité de notre industrie aluminium et renforcer notre souveraineté ?

Nous pouvons d’ailleurs être fiers et de la filière française, qui représente 10 % de la production européenne, et de compter sur notre territoire le premier site européen d’aluminium primaire : Aluminium Dunkerque. Dunkerque. La politique française de soutien à la filière a permis de développer ses capacités de production sur le territoire national, ce qui devrait permettre de couvrir 70 % de nos besoins actuels dès 2025.

Sur ce point précis du recyclage, nous devons, autant que possible, recycler les déchets à proximité de l’endroit où ils sont produits tant pour réindustrialiser la France que pour décarboner son industrie.

Ensuite, concernant la concurrence internationale accrue qui pèse sur cette filière, les droits de douane de 25 % annoncés par Donald Trump sonnent comme une alarme. La France plaide, comment elle l’avait fait lorsque des mesures similaires avaient été prises en 2018, pour un message de fermeté en matière de politique commerciale. L’Union européenne doit se départir de toute naïveté

nationale le 7 novembre 2024 vise à répondre à un besoin légitime de régulation du marché locatif des logements. Toutefois, en modifiant le régime fiscal des chambres d’hôtes

Contrairement aux meublés de tourisme, les chambres d’hôtes proposent des nuits uniquement avec des services associés, tels que le petit déjeuner, le ménage ou encore le linge de maison. Il s’agit d’une activité proche de la para hôtellerie, encadrée par des règles strictes, et n’ayant aucune incidence sur le parc immobilier résidentiel. Or, en alignant leur régime fiscal sur celui des meublés de tourisme, avec une réduction drastique de l’abattement fiscal à 50 % pour les chambres d’hôtes, contre 71 % précédemment, et une baisse significative du seuil de revenus à 77 700 euros, contre 188 700 euros auparavant, cette réforme menace la viabilité économique de nombreux exploitants. Cette activité procure des revenus limités, malgré une implication quotidienne importante et des horaires étendus, nécessaires pour maintenir le confort et la satisfaction d’une clientèle qui contribue aussi à l’attractivité touristique et économique de nos régions. Les exploitants de ces hébergements, souvent investis en milieu rural et engagés dans la réhabilitation de bâtiments anciens, jouent un rôle clé dans le soutien de l’économie locale et du tourisme de passage. Madame la ministre, cet alignement fiscal pourrait il être revu pour tenir compte des spécificités des chambres d’hôtes, dont le fonctionnement et les retombées sont radicalement différents de ceux des meublés de tourisme ?

Conformément au 2° du 1. de cet article 50 0, modifié par le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire, la location de chambres d’hôtes relève désormais du régime micro BIC dans la limite de 77 700 euros de chiffre d’affaires, avec un abattement de 50 %. Ce seuil est très supérieur à celui des locations meublées de tourisme non classées, qui a été abaissé à 15 000 euros, avec un abattement de seulement 30 %. Le législateur a souhaité maintenir un abattement différencié au bénéfice des meublés classés de tourisme et des chambres d’hôtes, incitant les propriétaires à se tourner vers un bien classé plutôt que vers des locations meublées de tourisme non classées. À cet égard, un seuil de 77 700 euros de chiffre d’affaires a paru au législateur suffisamment élevé pour tenir compte de la situation des petits propriétaires de chambres d’hôtes recherchant un revenu d’appoint. Par ailleurs, les propriétaires qui supportent des charges d’un montant supérieur à l’abattement de 50 % conservent la possibilité d’opter pour le régime réel, c’est à dire la déduction du montant réel En effet, le régime micro BIC est un régime d’imposition simplifié qui ne revêt aucun caractère incitatif et qui n’a donc pas pour vocation à offrir aux propriétaires une réduction de leur base imposable déconnectée des charges qu’ils supportent effectivement. Enfin, je vous précise que les nouvelles dispositions de l’article 50 du CGI, qui s’appliquent de plein droit aux revenus perçus à compter du 1 janvier 2025, n’appellent aucun décret pour leur application. La parole est à Mme Agnès Canayer,

En Seine Maritime, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a été créée le 1 janvier 2019 et s’est engagée dans cette procédure. En octobre 2023, par délibération, elle a mis en place le lissage des taux de Teom sur une durée de

Avec mes collègues parlementaires, nous avions interrogé à plusieurs reprises le ministre de l’économie et des finances, afin qu’il clarifie la situation. Nous sommes toujours sans réponse à ce jour. Aussi, madame la ministre, je vous pose deux questions, qui exigent des réponses claires. Premièrement, peut on appliquer des durées de lissage différentes en fonction des communes

Toutefois, il peut créer des zones de perception sur lesquelles sont appliqués des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu, c’est à dire des conditions de réalisation du service et de son coût. En l’occurrence, les zones créées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole doivent être justifiées au regard des éléments liés à la réalisation du service rendu et ne peuvent simplement correspondre aux différences de taux entre les communes avant fusion. Par ailleurs, lorsque des EPCI fusionnent, des règles particulières peuvent s’appliquer. Tout d’abord, lorsqu’un nouvel EPCI, issu d’une fusion, décide de ne pas délibérer immédiatement pour instituer la Teom, comme ce fut le cas pour Le Havre Seine Métropole en 2019, ce sont les délibérations antérieures qui continuent de s’appliquer.

Un dispositif d’unification progressive des taux d’une durée maximale de dix ans est alors applicable, sous réserve que des mécanismes différents de financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers préexistent au sein du groupement ou que l’unification des taux au sein de l’EPCI conduise à des hausses de cotisations pour les redevables. Ainsi, dans le cas du Havre Seine Métropole, le conseil délibérant a décidé de lisser les taux sur une période de quatre ans à compter de 2024. Durant cette période, l’intercommunalité détermine librement les modalités de l’harmonisation progressive des taux sous réserve de parvenir, à l’issue de la période de lissage, au taux cible de Teom dans chacune des zones qu’elle a définies. Cette période pourra être prolongée sur délibération de l’EPCI, sans que la durée totale de lissage puisse excéder dix ans.

et même nos villages. Les rodéos urbains peuvent être à l’origine de drames ; le département de l’Oise ne le sait que trop bien. Pour lutter contre ce fléau, la commune de Compiègne s’est démarquée en renforçant les effectifs de la police municipale et en intensifiant la vidéoprotection. Elle a ainsi récupéré depuis 2020 plus d’une cinquantaine de deux roues, souvent abandonnés par leurs propriétaires dans leur fuite. Malheureusement, madame la ministre, ces efforts pour mettre fin à de telles atteintes à la tranquillité publique ne sauraient être efficaces sans un appui et un accompagnement adéquats de l’État. Le maire de Compiègne, Philippe Marini, n’a pas de baguette magique. Plus que jamais, il a besoin du soutien du Gouvernement. Gouvernement. Pour aller plus loin, la commune de Compiègne se propose d’être ville expérimentale en matière d’utilisation des drones par la police municipale, ainsi que de recours au spray et au paintball de peinture codée. Puisque ces expériences ne peuvent avoir lieu sans réquisition du procureur de la République, je ne peux qu’appuyer la demande du maire de Compiègne, M. Marini, et vous demander d’y répondre favorablement. Je suis intimement convaincu que la mise en œuvre de ces mesures permettrait d’améliorer l’efficacité des agents de la police municipale et donc de

Madame la ministre, nous avons un choix à faire : laisser les maires seuls face à ce fléau ou leur donner enfin les moyens d’agir. Quelles mesures concrètes l’État compte t il mettre en place pour appuyer les communes dans cette lutte ? La parole est à Mme la ministre déléguée.

La lutte contre ce fléau s’intègre aux stratégies de partenariat et de réappropriation de la voie publique, qui sont au cœur de la restauration de la sécurité du quotidien. C’est le cas notamment à Compiègne, où les policiers agissent en prévention et de manière dissuasive par les opérations de voie publique que vous avez rappelées : quatorze opérations anti rodéos y ont été organisées par la police nationale en 2024. En partenariat avec les bailleurs, un travail est également mené pour identifier les lieux de stockage des engins. Enfin, des procédures judiciaires sont engagées, chaque fois que des éléments le permettent, avec l’aide du système de vidéoprotection de la ville.

L’exemple de Compiègne doit inspirer d’autres villes, qui doivent s’impliquer plus et mieux dans cette lutte. Même si le phénomène est loin d’être éradiqué, des résultats sont obtenus. En 2024, à Compiègne, la police nationale a procédé à six interpellations et engagé sept procédures judiciaires.

chemins régulièrement fréquentés, stations essence où se réapprovisionnent les conducteurs de deux roues – et les moments – mercredis et week ends – propices aux rodéos. Cette action ciblée a permis de saisir vingt six engins en 2024. mentionné l’emploi de sprays de produits de marquage codés (PMC). Cette approche a été expérimentée entre 2021 et 2023, notamment dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre, pour identifier les auteurs de dégradations. s’étant révélée peu conclusive, elle a été abandonnée. Appliqué aux rodéos urbains, en dehors des cas de flagrance, ce dispositif ne constituerait pas une preuve suffisante. Le Beauvau des polices municipales mené par le ministre François Noël Buffet offrira l’occasion de nous interroger de nouveau sur ces différents sujets. Le Gouvernement est fermement engagé pour offrir aux policiers municipaux les moyens d’agir efficacement pour répondre aux attentes croissantes des Français, dans le respect des principes constitutionnels et des prérogatives de l’autorité judiciaire.

mais le sujet évoqué semble prendre une tournure interministérielle. Cette question concerne tous les agents qui ont été exposés à l’amiante durant leur vie professionnelle ; je leur avais déjà consacré une première question orale, le 5 décembre 2023.

L’évolution statutaire de certains établissements du ministère des armées et les différents détachements, mises à disposition, mises en disponibilité et mises hors cadre qui se sont ensuivis, ont créé au fil du temps des injustices quant à l’ouverture de ces droits. Ces injustices ont été partiellement corrigées, pour les anciens ouvriers d’État, par la parution d’un décret rectificatif spécifique. Toutefois, il reste encore un certain nombre de personnels sous statut, fonctionnaires ou contractuels,

bénéficient de la cessation anticipée d’activité quand leurs fonctions professionnelles les ont exposés à l’amiante. Comme vous le savez, par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d’État a étendu ce dispositif aux anciens ouvriers de l’État qui n’étaient plus agents publics quand ils ont fait leur demande. Cette décision du Conseil d’État a conduit à une modification de la réglementation en 2022. Depuis cette date, il existe donc bien une différence selon le statut des personnes concernées. Les anciens ouvriers de l’État peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante. Mais tel n’est pas encore le cas des anciens fonctionnaires et des anciens contractuels de droit public qui ne possèdent plus la qualité d’agent public au moment de leur demande. C’est la situation

Une disposition législative étant nécessaire, elle a été inscrite dans la loi de finances initiale pour 2025. Je vous confirme que l’ensemble des ministères concernés travaillent de concert pour préparer le décret d’application afférent, indispensable pour rendre opératoire le dispositif. publié très prochainement pour qu’enfin tous les agents et les anciens agents qui ont été exposés à l’amiante au cours de leur carrière publique puissent bénéficier de la reconnaissance qui leur est due. La parole est à Mme Agnès Evren, ministre de l’intérieur. Madame la ministre, depuis plusieurs mois, la France enchaîne les tragédies : Thomas à Crépol, Matisse à Châteauroux, et maintenant Philippine, Élias et Louise à Paris, tous ces jeunes ont eu leur vie arrachée à coups de couteau par des barbares. Les coupables doivent être sévèrement punis et les élus doivent tourner la page d’un déni inadmissible. Le dernier rapport disponible de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) dénombrait, en 2020, 120 attaques au couteau par jour en France. Je répète : 120 attaques au couteau par jour ! À ce niveau, ce sont non plus des faits divers, mais bel et bien des faits de société qui touchent nos enfants. Élue à Paris, dans le XV arrondissement, je constate que notre ville fait face à une explosion de la violence. Coup sur coup, nous avons vécu

Les attaques au couteau se multiplient, mais quelle est sa réponse, à part le déni ? Arme t elle sa police municipale ? Non ! Massifie t elle le recours aux caméras et aux systèmes de vidéoprotection ? Non ! La réponse d’Anne Hidalgo et de la gauche parisienne est de distribuer des dépliants intitulés : « Porter un couteau, c’est se mettre en danger,

Les attaques commises au moyen d’une arme blanche ou de toute autre arme témoignent d’une violence qui atteint un niveau alarmant, d’un ensauvagement qui questionne profondément notre modèle de société et sa cohésion. Nous avons besoin d’un continuum de sécurité. Au delà des attaques dues au terrorisme ou liées à des pathologies psychiatriques, la prégnance du phénomène sur le territoire national commande d’y consacrer tous les moyens nécessaires pour y faire face. Mais l’aisance à se procurer un couteau et à le dissimuler rend très difficile la détection de ces armes par les forces de sécurité

La réponse est aussi interministérielle. Comme vous le savez, dans sa circulaire du 19 novembre dernier, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a demandé aux préfets d’élaborer des plans départementaux de restauration de la sécurité du quotidien. Plus de liberté d’action pour plus de résultats, voilà quel doit être le leitmotiv de ces plans mobilisant l’ensemble des acteurs du continuum de sécurité. Lutter contre les violences à l’arme blanche passe aussi, naturellement, par une réponse pénale à la fois efficace et sévère ; le garde des sceaux s’y emploie. Dès le premier écart grave, dès qu’il y a une menace, dès qu’il y a une gravité dans l’infraction, alors il doit y avoir une sanction.

question des statistiques, le phénomène n’est pas simple à quantifier. Je peux cependant vous indiquer qu’au sein de l’agglomération parisienne, les vols commis avec arme blanche ont reculé de 22 % entre 2023 et 2024. enfin à souligner le rôle que peuvent jouer les systèmes de vidéoprotection pour une intervention rapide et une prompte interpellation des auteurs de ces actes. Ce fut notamment le cas pour l’assassin de la jeune Louise. Madame la sénatrice, je peux vous assurer que nos policiers et nos gendarmes continueront d’agir sans relâche sur le terrain pour garantir la sécurité de tous les Français.

Ce site a refait parler de lui à la fin de 2024, avec la diffusion du documentaire intitulé. La population continue de s’interroger quant aux niveaux de pollution et de contamination radioactives des sols et des nappes phréatiques.

Un suivi hydrogéologique est pratiqué depuis 2023, mais uniquement sur la zone périphérique du site. L’État ne peut donc pas garantir l’absence de pollutions. Les nappes phréatiques voisines alimentent en eau potable la population de la majeure partie de l’agglomération de Reims ; il est donc impératif de connaître l’état sanitaire des sols et du sous sol. De plus, l’État n’a jamais évoqué l’opportunité d’une dépollution du site, privilégiant le scénario du silence et du déni, alors que le site est fermé depuis douze ans.

De 1957 à 2013, le CEA n’a fait qu’y réaliser des expériences de détonique pour observer la mécanique des explosions. Ces expériences se sont révélées utiles à la mise au point des armes de la dissuasion française, de réactions de fission ou de fusion nucléaire. Le CEA a cessé ses expériences sur le site de Moronvilliers dès 2013. Le site est alors entré dans une phase de remise en état général, sous le contrôle du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection qu’il n’y ait aucun impact sur la population ou sur l’environnement, à court comme à long terme. Des simulations sont réalisées sur cinq cents ans. Les travaux engagés sont compatibles avec les usages envisagés de cette friche industrielle ; ils se poursuivront durant les trois prochaines décennies.

hydrogéologique instauré en 2023 sur la zone périphérique du site fait apparaître des concentrations en uranium dans les eaux prélevées quarante fois inférieures à la valeur maximale réglementaire française pour les eaux destinées à la consommation humaine. Tout ce travail est fait en transparence, avec les élus locaux. Une commission locale d’information a été créée le 3 février 2017. Elle se réunit annuellement sous la présidence du sous préfet de Reims et rassemble les élus locaux. Les résultats des mesures effectuées dans les exutoires naturels et les eaux superficielles sont transmis par courrier à la fois à la préfecture de la Marne et à l’ensemble des maires concernés. Vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement est pleinement mobilisé, comme vous le demandez, pour assurer la transparence des informations et le suivi rigoureux de la situation environnementale du site.

nos policiers municipaux sont bloqués à l’âge du papier quand il s’agit de dresser des contraventions locales. Quel est le responsable de cette situation absurde ? Notre code de procédure pénale, qui n’a pas fait sa mise à jour « 2.0 Nos lois et règlements interdisent en effet d’avoir recours à une procédure informatisée pour des infractions à des arrêtés municipaux pris au titre des pouvoirs de police du maire. Nous prônons tous ici l’efficacité du service public. Dès lors, comment peut on accepter que nos élus locaux et nos policiers municipaux perdent un temps précieux à rédiger à la main des PV et les rapports qui les accompagnent ? Mais ce n’est pas tout ! Le même code impose que ces contraventions soient adressées à l’officier du ministère public pour qu’il apprécie l’opportunité des poursuites. Dans la pratique, ce dernier est débordé et finit généralement par les classer sans suite. Les conséquences sont bien réelles : perte de motivation de nos agents et de nos élus municipaux ; perte de confiance de nos concitoyens dans leurs institutions ; enfin, renforcement du sentiment d’impunité des fauteurs de troubles, ce qui peut les amener à récidiver ou à commettre des infractions plus graves.

des arrêtés de police des maires. Cette violation est réprimée par l’article R. 610 5 du code pénal. L’article R. 48 1 du code de procédure pénale, quant à lui, dresse une liste des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Cette liste ne comprend pas l’ensemble des infractions constituées par la violation des arrêtés de police du maire. En effet, ces infractions sont susceptibles d’être constituées dans des hypothèses extrêmement variées. Elles ne sauraient d’ailleurs être facilement traitées dans les bases informatiques du ministère de la justice. En outre, une telle forfaitisation n’apparaît pas nécessaire pour assurer une répression efficace en la matière. du décret du 15 février 2022, le non respect des arrêtés de police du maire est constitutif d’une contravention de deuxième classe et non plus simplement d’une contravention de première classe.

Vous nous dites que le Gouvernement est mobilisé aux côtés des élus ; je veux bien l’entendre. Il faut que les choses soient bien claires et que les élus puissent, demain, assumer leurs fonctions en toute sérénité. La parole est à Mme Valérie Boyer,

Arrêté dans la foulée, il est incarcéré à la prison des Baumettes, à Marseille. Le 1 octobre, le jeune homme écrit à ses parents ; il reste optimiste sur la suite de cette affaire. Malheureusement, trois jours après, et son enfer débute. Selon un document relaté par la presse, il a exprimé, à plusieurs reprises, ses craintes à l’encontre de son codétenu. En effet, il a lancé l’alerte trois fois par lettre, sans compter les appels à l’interphone. Arrive alors la soirée du 9 octobre, où le bruit d’une violence inouïe retentit dans la cellule. Son bourreau s’est servi d’un bol cassé pour le tuer, jusqu’à pratiquement le décapiter. Il lui a écrasé le visage. Comble de l’horreur, le meurtrier indique également avoir manipulé le corps de sa victime pour accélérer l’hémorragie. Ses parents ont appris les circonstances de la mort de Robin dans la presse. Je veux leur témoigner toute ma compassion. Au delà de sa famille, je crois que les Français attendent des réponses. Nous sommes tous dans la stupeur, le chagrin et l’incompréhension. Aussi, madame la ministre, même si je devine que vous allez me répondre qu’il ne vous appartient pas de commenter une affaire en cours, je vous demande de faire preuve de transparence sur ce drame.

qu’en janvier, dans les Yvelines, un individu condamné pour le viol de sa nièce mineure a été remis en liberté faute de date disponible pour son procès, bref – la liste est trop longue, hélas ! –, alors que bien des personnes dangereuses sont en liberté, pourquoi ce jeune homme, qui n’était pas dangereux, qui n’avait pas de casier judiciaire, qui avait un travail

au delà de six années scolaires consécutives – cette durée peut, par dérogation exceptionnelle, être allongée à neuf années scolaires consécutives. Pour nombre de fonctionnaires de l’éducation nationale qui ont obtenu un nouveau poste à l’étranger en 2019, la période de détachement va donc arriver à terme

alors que l’éducation nationale fait face à une crise de recrutement et que les rectorats découragent les détachements à l’étranger afin de limiter les pénuries de personnel dans l’Hexagone.

au Gouvernement de revenir sur cette limitation à six ans du détachement, au profit des reconductions tacites qui prévalaient auparavant. Ainsi, tous les enseignants détachés qui le souhaitent

heures. Des formations départementales et académiques sont accessibles sur tout le territoire, avec des modules nationaux consacrés à leur métier ou partagés avec les professeurs.

En parallèle, ces derniers peuvent compter sur l’accompagnement des professeurs ressources du service de l’école inclusive et des conseillers pédagogiques des établissements. Dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, un professeur ressource sera affecté dans chaque département d’ici à 2027, en complément des spécialistes de l’autisme déjà déployés. Depuis la rentrée 2024, nous expérimentons les pôles d’appui à la scolarité (PAS) dans quatre départements. Ces pôles, qui associent éducation nationale et secteur médico social, interviennent dès le plus jeune âge et sur tous les temps de l’enfant : scolaire, périscolaire, extrascolaire. Dès 2025, plus de 200 PAS supplémentaires seront implantés pour mieux répondre aux besoins

de la recherche. Monsieur le ministre, depuis la loi du 27 mai 2024, l’État est désormais compétent pour la prise en charge financière des accompagnants d’élèves en situation de handicap durant la pause méridienne. C’est au rectorat qu’il appartient de définir les modalités de cet accompagnement humain. Cette loi répond à un besoin évident de solidarité nationale à l’égard des familles. Néanmoins, sa mise en œuvre est source de gros problèmes au quotidien dans les écoles. Plusieurs communes du Calvados sont confrontées à ces

Pour cela, nous nous appuyons sur une analyse fine des besoins de chaque élève, en prenant en compte les recommandations des MDPH et l’expertise des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) ou des pôles d’appui à la scolarité.

Enfin, nous avons fait le choix d’un déploiement renforcé des pôles d’appui à la scolarité pour apporter aux familles des réponses rapides et adaptées : premièrement, des aménagements pédagogiques éducatifs adaptés ; deuxièmement, la mise à disposition de matériel pédagogique spécifique ; troisièmement, un accompagnement renforcé par des professionnels de l’éducation nationale et du secteur médico social. Notre objectif est simple : garantir à chaque élève les meilleures solutions, sans que les familles aient à naviguer seules dans des démarches administratives complexes. Madame la sénatrice, soyez assurée de notre engagement à faire de l’école inclusive une réalité. La parole est à Mme Sylviane Noël,

et 140 000 traumatismes par an, dont une grande part est prise en charge par les médecins de montagne. Ces cas de traumatologie sont souvent graves et nécessitent une réactivité et une technicité qui se passeraient d’obstacles administratifs et financiers. nationale de l’assurance maladie (Cnam) impose notamment aux médecins de montagne un recours systématique au centre 15 pour administrer des antalgiques intraveineux comme la morphine. Par ailleurs, l’acte visant la prise en charge d’une urgence traumatique, neurologique, respiratoire ou cardiaque ne peut être coté que si le patient est adressé ensuite aux urgences. Pour nos médecins de montagne, cette mesure est inadaptée aux réalités de terrain où, en cas de fracture ou de luxation sévère, chaque minute compte. Ces délais supplémentaires mettent directement en danger la vie des patients. En outre, les actes d’urgence et de traumatologie, pourtant essentiels, ne sont pas valorisés à la hauteur des coûts spécifiques qu’ils engendrent en zone de montagne. Ce problème a été aggravé par la modification des majorations MN, MM, et des modalités d’application des cotations de week end et de garde type F et CRD, applicables depuis le 22 décembre 2024. Ces majorations, désormais limitées aux seules consultations régulées par le 15 ou aux urgences vitales, entraînent une perte de rémunération significative pour les médecins, qui, durant toute la saison et au delà, sont mobilisés la nuit, le week end et les jours fériés. Ces contraintes menacent directement la pérennité de l’offre de soins en Haute Savoie, où les coûts d’exercice en montagne sont bien supérieurs à ceux que l’on rencontre en milieu urbain. En outre, il ne faut pas oublier la forte attractivité de la Suisse voisine pour ces personnels. à des ajustements, les fermetures de cabinet risquent de se multiplier, d’aggraver la désertification médicale et de reporter la charge sur des hôpitaux déjà bien saturés. Je souhaite donc connaître les mesures concrètes envisagées par le Gouvernement pour alléger ces contraintes

La convention médicale signée en juin 2024 résulte de discussions riches entre l’assurance maladie et les représentants des médecins libéraux, l’objectif premier étant d’améliorer l’accès aux soins. aux soins. Les soins non programmés ont fait l’objet d’une réorganisation, laquelle était nécessaire, pour éviter les dérives tarifaires et pour préserver les ressources médicales dans nos territoires. Désormais, la régulation par le service d’accès aux soins et la permanence des soins ambulatoires permet de mieux mobiliser les ressources là où elles sont indispensables. La convention rappelle ainsi que les cotations d’urgence non régulées doivent rester exceptionnelles et être réservées aux cas justifiant une hospitalisation. Afin d’accompagner cette transition sans déstabiliser les acteurs, le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins a demandé à l’assurance maladie et aux agences régionales de santé de privilégier la pédagogie. concerne les cabinets de montage, le ministre est particulièrement attentif à leurs spécificités. Depuis 2015, le dispositif de labellisation en Auvergne Rhône Alpes a permis de financer cinquante quatre cabinets pour un peu plus de 2 millions d’euros. De plus, la nomenclature prévoit déjà un supplément pour les examens radiologiques effectués en montagne.

aménager le territoire, à permettre à chacun de construire son développement, tout en assurant la cohérence et la cohésion de la Nation ! Belle gageure ! Pour ce faire, les gouvernements ont mis en place des dispositifs perlés, à l’instar, dernièrement, des pactes territoriaux, qui fonctionnent plus ou moins.

Face à une telle situation et à ce déferlement d’indicateurs, les élus ont élaboré, avec l’État et le département, une stratégie pour l’avenir du Cambrésis 2027. Le préfet Lalande l’a cosignée en 2019. Depuis : rien Ma question est donc simple, madame la ministre : allez vous honorer la parole de l’État ? Allez vous permettre au Cambrésis d’accéder à un développement équitable et équilibré ? La parole

Je pense aussi au programme France Ruralités : six communes rurales bénéficient du programme Villages d’avenir. Enfin, l’État intensifie aussi dans le Cambrésis, comme partout, ses efforts dans la lutte contre les violences intrafamiliales

Le but était de recréer du lien, de la sociabilité, en mobilisant et en impliquant nos villages. Cette belle opération visait à redonner de l’âme à nos petites communes autour d’un café. Cinq ans plus tard, le bilan est plus que mitigé, en particulier dans le département des Ardennes. Sur les 1 000 cafés

La déception n’est pas que d’ordre statistique ou comptable. Si, dans certaines situations, des projets n’ont pu aboutir, dans d’autres cas, des communes se sont heurtées à des retraits soudains et inopinés de la part d’opérateurs pas toujours scrupuleux, voire à des pressions injustifiées sur les gérants. C’est le cas dans trois communes de mon département. Alors qu’elles avaient financé, soutenu et facilité ces projets en utilisant tous les instruments disponibles qu’une commune peut mettre en œuvre, elles se heurtent à des retraits sauvages de la part de gérants sans scrupules, qui n’ont parfois investi aucun euro préalablement. préalablement. De ces cafés promis, elles ne voient, si je puis dire, ni la couleur ni l’odeur. Elles font face ensuite à des difficultés financières. Madame la ministre, comment aider ces communes qui ont été victimes de démarches aux limites de la malveillance, dire de la malhonnêteté dans certains cas ? Comment les aider à poursuivre des projets dans lesquels elles se sont tant impliquées et pour lesquels elles ont beaucoup donné ? Comment garantir un objectif qui réside dans le nom même de l’opération : « 1 000 cafés » ? Je ne voudrais pas conclure comme on l’a fait à propos de Louis XV : « France, ton café fout le camp

trimestriel ou semestriel, assuré et stable, ces entreprises réalisent des prestations de sous location de courte et moyenne durée. Souvent proposées des plateformes en ligne, ces offres s’adressent, en majorité, à une clientèle touristique. Ce nouveau procédé réduit mécaniquement l’offre de logements permanents disponibles pour la population locale. Alors que la France pâtit d’un fort manque de logements, cette situation négative ne fait qu’accentuer le déséquilibre entre l’offre et la demande. de noter également que ces contrats de sous location sont moins encadrés d’un point de vue juridique pour les sous locataires, qui ne bénéficient pas des mêmes garanties que les locataires. En outre, la sous location ne relève pas d’un régime fiscal plus avantageux que la location. Ce développement dérégulé de la sous location participe à une sorte d’ubérisation de la gestion locative dans ce pays. Par exemple, dans le Briançonnais, dans mon département, les prix du logement empêchent les locaux et les travailleurs saisonniers de se loger. Je parle non pas d’acquisition foncière, mais simplement de location.

La procédure de déclaration et d’enregistrement en mairie est aujourd’hui généralisée. Les fausses déclarations et le non respect par la plateforme d’une injonction

délimiter dans leur plan d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. Elles peuvent aussi limiter à quatre vingt dix jours par an la durée de location de résidences au lieu de cent vingt jours auparavant une sanction en cas de dépassement. Enfin, le régime fiscal des meublés touristiques a été rapproché de celui de la location nue. Ces premiers éléments sont, je pense, de nature

par plusieurs centaines de jeunes qui n’ont pas été reconnus mineurs et qui contestent cette décision auprès du juge des enfants. Cette occupation d’un lieu culturel dure depuis maintenant plus de deux mois. Il faut absolument sortir de cette impasse. La situation devient d’autant plus alarmante que nous constatons l’impuissance des pouvoirs publics à faire face à une détresse bien réelle et l’absence d’actions concrètes de l’État, dont la responsabilité

Les jeunes qui sont reconnus mineurs sont évidemment pris en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l’enfance, mais les autres se retrouvent à la rue la plupart du temps, sans ressource ni perspective. La Ville de Paris ne peut pas remplir seule une mission dont la responsabilité incombe à l’État, mais elle est prête à l’accompagner comme elle l’a toujours fait. Avec plusieurs sénatrices et sénateurs de Paris, nous avons d’ailleurs écrit au Premier ministre il y a quelques semaines à ce sujet, mais nous n’avons

dont 46 800 rien qu’à Paris. Cela représente en dépenses pour l’État, monsieur le sénateur, pour la seule Île de France, un budget de 1,6 milliard d’euros. L’État est donc particulièrement et pleinement engagé

Si ce recours n’est pas favorable, ces personnes seront alors en situation irrégulière et devront, conformément à la loi, quitter le territoire. Pour accompagner Pour accompagner la collectivité de Paris dans sa mission de prise en charge, l’État a répondu très présent. En novembre 2024, la préfecture de police a signé avec la Ville de Paris une convention pour l’appui à l’évaluation de la situation,

En Bretagne, les mytiliculteurs font face à des difficultés croissantes liées à l’augmentation de la prédation. Les oiseaux, les daurades et les araignées de mer s’attaquent aux moules dans les baies mytilicoles bretonnes. Si les Côtes d’Armor sont particulièrement touchées,

les moyens de lutte contre cette prédation présentent des limites et ne sont donc pas pleinement efficaces. Le cadre réglementaire apparaît inadapté aujourd’hui, dans la mesure où la mytiliculture ne dispose d’aucun instrument, hors pêches expérimentales, pour réguler les espèces

l’Union européenne, la région Bretagne et les collectivités territoriales apportent des aides, mais elles ne peuvent être débloquées que pour des opérations collectives et ne couvrent aucunement l’ensemble des dépenses engagées par les producteurs. C’est pourquoi, madame la ministre, le Gouvernement doit réagir avant le mois d’avril, qui marque le début de la période de prédation par l’araignée de mer. Allez vous faire évoluer d’ici là le cadre réglementaire en vue d’autoriser les effarouchements dans les concessions de cultures marines et d’avancer sur le statut de prédateur ? Allez vous également prévoir un volet assurantiel afin que l’État améliore son soutien à la filière mytilicultrice et aille au delà des aides dites, qui n’ont toujours pas été perçues

leur santé économique. Un certain nombre d’outils existent, comme le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa). Il permet de financer l’équipement matériel pour lutter contre les prédations et contribue au fonds de mutualisation aquacole. Un dispositif de garantie est également prévu en cas de contractualisation avec une compagnie assurantielle privée, pour répondre à votre question sur l’assurance. Ce fonds de mutualisation doit être constitué par les professionnels, qui ont la main sur sa structuration et sur son fonctionnement, ainsi que sur la définition des risques à couvrir. L’État se tient prêt à apporter tout le soutien nécessaire à l’établissement de ce fonds.

assez inattendues – de la Commission européenne visant à instaurer des moratoires de chasse ou des réductions significatives des prélèvements pour certaines espèces d’anatidés comme le canard souchet, le canard pilet, le canard siffleur et le fuligule milouin. Quelle est la position du Gouvernement sur ces annonces européennes

En effet, les estimations actuelles des populations d’oiseaux migrateurs reposent en grande partie sur des données géographiques restreintes, excluant notamment des zones essentielles comme la Sibérie, qui constitue un habitat majeur pour ces espèces. ces espèces. Les chasses au gibier d’eau réalisées dans le cadre de plans de gestion adaptative sont un levier de préservation des espèces, contribuant à une collecte précieuse de données pour affiner notre connaissance des dynamiques dynamiques migratoires. Quelles démarches le Gouvernement entend il engager auprès des instances européennes pour garantir la fiabilité et l’exhaustivité des données prises en compte dans les décisions de gestion des espèces migratrices ? Vous devez défendre la mise en œuvre d’une gestion adaptative reposant sur des partenariats solides avec les acteurs locaux,

Le ministère examine actuellement les mesures que la France pourrait mettre en place pour y répondre. Le Gouvernement plaide pour une prise en compte rigoureuse des données scientifiques disponibles, en particulier de celles qui sont fournies par le terrain sur la population. Il est attentif aux impacts sociaux et culturels que vous évoquez. Bref, le Gouvernement souhaite défendre une approche équilibrée et concertée de la chasse, ce qui nécessite de garantir la conservation des espèces tout en permettant une pratique durable et responsable des activités de chasse. La parole

La prévention sur les dangers de l’inhalation du protoxyde d’azote et les restrictions à la vente de cartouches doivent incontestablement être renforcées. En parallèle, d’autres dispositions sont nécessaires pour réduire l’impact environnemental et financier du traitement Plusieurs solutions sont envisageables. Une première consisterait à obtenir des industriels la modification des valves d’étanchéité des contenants afin de prévenir toute explosion. La deuxième serait d’instaurer une écocontribution sur les cartouches et bonbonnes, comme cela se fait pour d’autres types de déchets qui présentent des risques sanitaires et environnementaux élevés. La création d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pourrait enfin être étudiée, afin que les structures publiques, et donc les contribuables, n’aient plus à supporter financièrement les coûts de traitement de ces déchets.

Cette proposition nous semble pertinente, car il vaut mieux intégrer ces bouteilles et cartouches à une filière existante que d’en créer une nouvelle. Par ailleurs, la mise en place d’une soupape de sécurité sur les bouteilles